Ce le 1er ministre des dames et messieurs les ministres, mes chers collègues, la séance est ouverte, le compte rendu intégral de la séance du 27 juillet qui publié sur le site internet du Sénat : je n'ai pas reçu d'observation. Je n'en vois point. Avant de commencer les questions d'actualité au gouvernement, je voudrais rappeler que la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation pour le renforcement du dialogue social, a pu aboutir à un accord ce matin, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la confiance dans la vie politique est parvenu à l'adoption d'un texte commun, en revanche, il n'a pas été possible d'aboutir à un texte commun sur le projet de loi organique. Nous examinerons demain mercredi 2 août il y a noté pour vos agendas à 16 heures les conclusions des 2 commissions mixtes paritaires, qui ont abouti à un accord pour le projet de loi organique, le gouvernement a décidé une nouvelle lecture cette lecture sur proposition de la Commission et avec l'accord du gouvernement et j'6 de tous les groupes politiques aura lieu vendredi 4 août dans l'après-midi à 15 heures et éventuellement le soir. Je pense qu'il n'y a pas d'opposition, ça vous évitera une semaine complémentaires voilà et non en est ainsi décidé après cette large consultation démocratique de ma part. En conséquence. noté le délai limite de dépôt des amendements de séance sur le projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique pour être, c'est à l'ouverture de la discussion générale, la discussion générale-elle fixée à à une heure par l'opposition, il en est ainsi décidé. Par lettre en date du 28 juillet 2017, monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, m'a fait connaître qu'en application de l'article L aux 137 et nos 320 du code électoral, monsieur Laurent Dutheil est appelé à remplacer en qualité de sénateur du Val-de-Marne monsieur Luc Carvounas, à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, confirmant son élection à l'Assemblée nationale. Nous ne Nous ne souhaitons la bienvenue. Et son mandat a commencé samedi 29 juillet 2010 à 0. L'ordre L'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement, je vous rappelle que notre séance et retransmis sur le site internet du Sénat sur Public Sénat et sur Facebook,

Monsieur le président, ma question s'adresse au 1er ministre porte sur l'organisation à la préparation de la consultation de sortie de l'accord de nourrir monsieur le 1er ministre dans votre déclaration de politique générale, vous avez affirmé que l'État de jouer pleinement son rôle d'acteur et de garant du processus de l'accord de Nouméa. Vous en avez même fait. Un engagement personnel, je tiens à saluer ce volontarisme qui succède à l'attentisme et aux atermoiements du quinquennat précédent mais il faut passer de la parole aux actes, vous avez vous-même rappelé que s'il n'est pas saisi d'ici mes prochains par l'assemblée délibérante de Nouvelle-Calédonie, l'État devra organiser en novembre 2018 la consultation pour l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie, en clair, dans 15 mois la Calédonie décidera de son accession ou non à l'indépendance, alors que l'issue de ce référendum est connu d'avance, le risque est grand que ce scrutin de nature exagérément binaire mal préparée remette le feu aux poudres. Permettez-moi de rappeler ce que Michel Rocard affirmait. Personne ne peut avoir dans la tête que la question qui va être posée à ce référendum soient choisis de manière à diviser les Calédoniens en 2 paquets les égo, parce que là on est sûr qu'ils recommenceront à se taper dessus, monsieur le président du Sénat, vous avez vous-même affirmé à plusieurs reprises que l'État devait nous accompagner dans la recherche des convergences nécessaires à la définition de notre destin commun au plan local, nous avons pris l'initiative d'organiser les états généraux de l'avenir, forme de palabres, l'océanienne pour échanger et rechercher avec la population, l'ensemble des forces politiques, ce qui nous unis, ce qui nous ressemblent, ce qui nous rassemble, afin que cette consultation ne soit pas mortifère monsieur le 1er Ministre, êtes-vous prêt lors de votre venue annoncer en Nouvelle-Calédonie, donc je vous rappelle la devise de paroles, terre de partage à vous engager dans ce grand pas là pour l'avenir, et puisque vous avez insisté sur la dimension personnelle de votre engagement, pourriez-vous nous dire comment vous comptez traduire celui-ci dans les faits, monsieur le 1er ministre la parole de l'État est attendu à Nouméa, la parole de la France est attendu dans le Pacifique, je vous remercie. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, fragile, vous m'interrogez sur l'engagement du gouvernement et sur mon implication personnelle dans la construction de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, je vous en remercie, je veux vous dire à nouveau combien je suis conscient des enjeux et des défis considérables qui nous attendent collectivement en Nouvelle-Calédonie. Comme vous je veux éviter que les tensions s'avive à l'approche de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté. J'ai indiqué dans la déclaration de politique générale, quelle était l'ambition du gouvernement sur ce sujet, vous savez Monsieur le Sénateur que dès ma nomination, j'ai essayé de rencontrer toute une série d'acteurs politiques, parlementaires ou non et d'acteurs culturels de Nouvelle-Calédonie pour mieux saisir pour mieux mesurer et pour tout dire, pour mieux comprendre l'ampleur de ces défis et la complexité de ces enjeux, les faits Monsieur le Sénateur, et je vais continuer à le faire, comme l'ensemble du gouvernement d'ailleurs avec un esprit d'écoute et avec un esprit auquel vous êtes attaché, car c'est une valeur océanienne d'humidité, c'est l'esprit qui a guidé la visite de Madame la Ministre, en Nouvelle-Calédonie. Que je veux saluer à la effectué au cours de la semaine dernière son 1er déplacement dans les outre-mer, en choisissant de se rendre d'abord en Nouvelle-Calédonie pour y rencontrer. Elle aussi, pour mieux comprendre, mieux saisir mieux mesurer l'ensemble des acteurs du processus et au-delà. L'humilité que je crois indispensable pour aborder les questions qui sont devant nous, c'est d'abord une humilité devant la force de l'engagement de celles et ceux qui ont vrai parfois au prix de leur vie pour tracer un chemin de paix et marcher de concert vers ce destin commun qui est désormais un acquis. Et vous avez, Monsieur le Sénateur, je le sais, contribuent à ce chemin, notamment en proposant que le drapeau du FLNKS soit érigé à côté du drapeau français. Cette humilité, c'est aussi celle qui doit nous saisir, devant la responsabilité collective que nous avons, nous tous, c'est-à-dire les acteurs du processus de l'accord de Nouméa. Au fond, nous devons organiser dans la transparence, un scrutin dont la légitimité ne pourra pas être contesté, c'est une priorité de notre action, c'est une priorité de l'action et c'est une priorité, difficiles à atteindre techniquement, vous le savez. Et nous voulons aussi profiter des fruits de la réflexion souvent remarquables, menés par les nombreux experts missionnés par les nombreux gouvernements qui se sont, eux, intéressé à ce sujet, il y a de la connaissance acquise il y a de l'expérience acquise et il serait absurde, voire contre-productif de vouloir s'en passer, je vous dis ça, Monsieur le Sénateur, parce que l'ensemble du gouvernement entend s'inscrire dans une histoire et dans une continuité dans ce processus, c'est aussi une forme d'humilité mais je pense que cette indispensable. Nous avons et nous pouvons nous appuyer sur des acquis irréductibles, qui sont le Havre, je veux les citer, de l'amitié civile et de la réconciliation qui ont été engagés par Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur nous avons un grand nombre de points de convergences, qu'il s'agisse des valeurs aux sources de la société calédonienne comme de l'organisation institutionnelle ou encore du principe de la citoyenneté calédonienne, vous avez rappelé monsieur le sénateur, la devise de la Nouvelle-Calédonie, terre de paroles perdent de partage, vous souhaitez à juste titre, que l'État, plus encore que le gouvernement. Qui est à la fois acteur et arbitre du processus est lui aussi une parole, c'est le sens du déplacement de Madame la ministre, qui a insisté sur à l'occasion de son déplacement, l'enjeu de la jeunesse, la lutte contre l'insécurité, le soutien à la filière du nickel, la préservation de la biodiversité, j'aurai l'occasion, vous l'avez évoqué, monsieur le sénateur, de me rendre en Nouvelle-Calédonie, au cours de la première quinzaine du mois de décembre, après que les échéances électorales auront permis de renouveler les sénateurs de de de Nouvelle-Calédonie après aussi que nous aurons réuni au mois d'octobre, un comité des signataires pour justement et dans le détail, étudier les conditions d'organisation de la consultation qui se tiendra au mois qui se je voudrais profiter de ce moment pour dire Monsieur le Sénateur, que je compte bien que l'échange que nous aurons à l'occasion du comité des signataires qui sera précédée par beaucoup d'entretien puisque nous permettent d'échanger des bouts de paroles auxquelles l'ensemble des acteurs de Nouvelle-Calédonie sont eux attachés je voudrais aussi dire que se prononcer sur l'accession à la pleine souveraineté. ça n'est pas se prononcer pour ou contre le destin commun, le destin commun, il est acquis, il était un des acquis de l'ensemble des discussions de l'ensemble du partage, il y a eu depuis maintenant de nombreuses années il ne doit pas être remis en cause, je vous remercie, monsieur sanitaire. Merci monsieur le 1er ministre. La parole est maintenant notre collègue Madame Malherbe, le groupe du Rassemblement démocratique et social européen et pour 2 minutes. Merci monsieur le président, Mesdames et messieurs les Ministres, j'aurais pu à nouveau questionner le gouvernement sur la taxe d'habitation qui reste une préoccupation majeure des élus locaux mais je souhaitais évoquer un autre sujet d'inquiétude, qui concerne à la prévention des risques incendie monsieur ministre de l'Intérieur, récemment, le sud de la France et la Corse ont fait face à de violence, d'incendies qui ont réduit en cendres près de 4000 hectares de forêt, blessant au passage les pompiers et forces de l'ordre et secouristes, ils font preuve d'un très grand courage au péril de leur vie et je pense que nous pouvons tous ici leur rendre hommage, le 14 juillet dernier dans mon département des Pyrénées-Orientales au boulot et mort à cela, s'il y a près de la frontière espagnole, le feu a consumé 190 hectares et mobilisé plusieurs centaines de pompiers Monsieur le ministre ma question au-delà des outils que l'on peut donner aux pompiers et aux forces de sécurité pour lutter contre les incendies, concerne les moyens de prévention que l'on peut développer et valoriser parmi ces moyens, on peut rappeler ce qui concerne la défense des forêts contre les incendies, pour laquelle les départements et les communes devront en particulier avec l'entente de la forêt méditerranéenne, on peut aussi saluer les communes qui ont mis en place des réserves intercommunal de sécurité civile les risques dans les Pyrénées Orientales en particulier pour assurer une surveillance des massifs en lien avec les pompiers et l'ONF ainsi je souhaite insister tout particulièrement sur l'action des communes qui accompagne à l'installation d'éleveurs dans le cadre du Silvo pastoralisme ou qui accompagne les propriétaires de masse isolé dans le défrichement et l'entretien des espaces naturels. Par ailleurs, nous constatons qu'il existe des disparités d'une région à l'autre dans l'application de la réglementation en matière de prévention et parfois entre 2 communes d'un même département, ma question est simple, monsieur le Ministre, monsieur le Ministre, comment reconnaître et valoriser le rôle préventif joué par les communes rurales, y compris financièrement et aussi comment harmoniser la prévention sur l'ensemble du territoire national pour une plus grande efficacité. Merci pour vous répondre à la parole, déclare au ministre d'État, ministre de l'Intérieur que Gérard Collomb pour 2 minutes. Monsieur le président, ma mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices madame la sénatrice R Malines Malherbe. Je connais votre attention à la situation que nous venons de vivre et que nous vivons encore aujourd'hui. Nous étions la semaine dernière, d'abord en Corse, où près d'Olmetta quelque 1300 hectares de forêt ont brûlé, nous étions le lendemain avec Monsieur le 1er ministre à Bormes-les-Mimosas, où l'incendie était immense et où 12000 personnes ont dû être déplacés dans la nuit, je veux saluer, comme vous l'avez fait à cette occasion, le travail de toutes celles et de tous ceux qui se sont engagés. Le travail évidemment de nos sapeurs-pompiers de nos forces de protection civile qui était sur le terrain et croyez-moi, ils étaient profondément engagé la première action, comme vous l'avez dit, Madame la sénatrice, c'est la mort d'empêcher que le feu ne prennent, et donc d'avoir une autre vision de l'urbanisme et de la nature de ce que vous dites de l'entretien fait dans les zones agricoles, la 2ème c'est ensuite d'avoir les moyens disponibles et c'est pour cela qu'avec le gouvernement, malgré les difficultés financières, nous avons décidé de commander 6 avions nouveaux pour les prochaines années, de manière à avoir des moyens à la hauteur des difficultés qui peuvent être les nôtres. La parole est maintenant notre collègue Jean-Jacques Filleul, pour le groupe République en marche. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la ministre chargée des transports, ce dernier week-end de retours et départs des vacanciers a été marquée par une pagaille monstre à la gare Montparnasse, celle-ci ne pouvait plus exercer ses fonctions primaires accueillir les voyageurs et faire circuler les trains de nombreuses hypothèses ont été émises pendant ces 72 heures, en particulier sur la nature de la panne qui a bloqué des milliers de voyageurs et perturbé toutes les gares du réseau ouest Atlantique cette situation grave par sa longueur et les perturbations qu'elle a entraîné n'est pas admissible, le service public est profondément touché par cet preuve nous savons votre volonté, Madame la Ministre, vous êtes venu présenter votre feuille de route, le 20 juillet dernier devant notre commission Aménagement et Territoires et développement durable : votre projet est ambitieux, nous le soutenons SNCF réseau doit faire l'objet de lourds investissements pour rénover et moderniser l'infrastructure ferroviaire dans sa variété et sa multiplicité, il n'en reste pas moins que ces dysfonctionnements dont l'ampleur dépasse tous les incidents quotidiens du réseau sont inquiétants, d'autant que la concurrence voyageurs issu du 4ème paquet ferroviaire européen s'impose pour demain, c'est-à-dire le 2022 je veux rendre hommage à la sagesse des passagers en déficit d'informations alors patience ou fatalisme face à ces retards et suppressions de trains qu'elles ont subi et subissent encore aujourd'hui ce défaut d'information pas SNCF la longueur des recherches pour identifier l'origine de la panne ont entraîné des polémiques et surtout de nombreuses questions, madame la ministre, au vu de cette situation, comment avez-vous réagi, quelles sont vos exigences vis-à-vis de la SNCF et dans l'immédiat, quelles mesures envisagez-vous de prendre, je vous remercie.

Un signalement de défaut sur la basse tension du poste de qui contrôle la signalisation sur les 10 kilomètres de voies qui précède la gare Montparnasse. A été relevé par les équipes cette panne car il s'agit bien d'une panne a le double la double caractéristique d'être à la fois complexe à identifier car les stations dans lesquelles intervient la panne sont remplis de connecteurs il faut identifier le bon endroit où le collecteur ne fonctionne plus et d'être susceptibles de poser des risques graves à la sécurité des voyageurs car le défaut de basse tension peut avoir pour effet de faire passer un feu rouge, un feu Vert. Ce qui pose des questions de sécurité évidentes. La décision qui a été prise par la SNCF, a été donc d'essayer dans les meilleures conditions de rapidité d'identifier la panne. Mais elle s'est heurtée évidemment à la difficulté de l'identification de cette panne. à la difficulté de réorganiser le plan de transport sans savoir quand la panne serait identifié et résolu. Et à l'incroyable intensité du trafic dans ce week-end de chassé-croisé, et demi de passagers SNCF ce week-end 80000 70000 passagers impactés par la panne et 3500 passagers qui n'ont pas pu être acheminés la situation et cette situation n'était évidemment pas satisfaisante, vous le savez, je le sais, tous les Français l'ont compris et le président d'SNCF Mobilités comme le président d'SNCF réseau que j'ai reçu aujourd'hui avec madame la ministre des Transports. évidemment admis et en ont parfaitement conscience. Face à ces difficultés, monsieur le sénateur, et comme souvent dans les crises, nous avons vu des choses extrêmement insatisfaisante et d'autres qu'il faut souligner dans les choses insatisfaisant le temps passé pour identifier l'origine de la panne, la difficulté à mettre en place des process de travail en mode dégradé car certes, car certes. Vous voulez qu'on évoque les conditions dans lesquelles le le le le réseau a été régénérée pendant les 5 dernières années, monsieur le sénateur. Les 10 dernières années, les 15 dernières années. Monsieur le sénateur, il nous a fallu et il nous faudra et c'est le sens de l'intervention de Madame la Ministre, qui s'est rendu sur les lieux dès dimanche et qui est retourné le lundi,

j'ai parfaitement conscience du charme et de l'intérêt, et même de l'opportunité qui s'attache aux grands projets mais nous devons, pour des raisons de sécurité, il y a ici un certain nombre d'élus de territoire qui savent combien ces questions de sécurité sont importantes et qui ont des mauvais souvenirs. Pour des raisons de sécurité, pour des raisons d'efficacité, nous devrons consacrer des moyens à l'entretien des réseaux, c'est une priorité, c'est une priorité, et elle sera assumée. Un mot encore, Monsieur le Sénateur, pour ne pas être trop long pour dire que nous avons demandé au président de la SNCF, réseau et au président de la SNCF Mobilités de faire évidemment tout le retour d'expérience nécessaire sur untel incidents que ce soit dans la mobilisation dès gilets rouges qui permettent d'informer les utilisateurs, que ce soit dans la qualité ou en l'espèce, dans l'absence de qualité de l'information qui a été transmise aux usagers qui venaient de sources différentes et qui était donc souvent imprécise et parfois contradictoires, ce qui n'est pas acceptable, nous avons SNCF réseau SNCF Mobilités à des progrès considérables à faire, c'est le sens des remarques précises, claires et fermes que Madame la ministre des Transports et moi-même avons formulé aux responsables de l'entreprise, mais je voudrais aussi dire monsieur le sénateur, parce que ça n'empêche pas que nous ne soyons pas satisfait, je voudrais aussi dire qu'à l'occasion de cette crise et c'est au fond un bel aspect que nous devons souligner, nous avons aussi vu ça n'excuse pas la satisfaction mais nous avons aussi vu des personnels se mobiliser revenir de leurs vacances pour essayer de faire face à une crise qui était une crise pénible et difficile, nous avons aussi vu Monsieur le sénateur, des gens qui oeuvrait jusque tard la nuit parce qu'il fallait apporter un service à l'usager et je veux aussi aussi le souligner. La parole est maintenant. Collègues Laurence Cohen pour le groupe communiste républicain et citoyen pour 2 minutes. Merci monsieur le président, le 2 juillet dernier, le 1er ministre de présenter un plan intitulé garantir le droit d'asile, mieux maîtriser les flux migratoires, en réalité, il s'agit avant tout d'une politique dissuasive, tandis que les droits élémentaires des migrants continuent à être bafoués récemment 156 migrants, parmi lesquels des mineurs ont été arrêtés à la gare de et reconduit brutalement à la frontière franco-italienne par les forces de l'ordre ils essayaient juste de déposer une demande d'asile en toute légalité cette reconduite à la frontière est une violation des droits humains les plus fondamentaux, Cédric et cet agriculteur militant des droits humains, les accompagnaient et était lui aussi une nouvelle fois arrêté pour délit de solidarité, le rapport de l'organisation Human Wright Swatch sur les violences commises par les forces de police à Calais à l'encontre de 400 à 500 migrants est lui aussi accablant l'emploi du gaz poivré courant, nombreuses sont celles et ceux qui sont choqués, à juste titre par cette violence institutionnelle qui émane hélas du pays des droits de l'homme, le président de la République a affirmé que, d'ici la fin de l'année, il ne voulait plus personne dans les rues, dans les bois, vous avez vous-même annoncé, Monsieur le Ministre, la création de 200 d'accueil dans les routes de France et demandé un rapport sur les violences, ma question est donc simple pouvez-vous nous préciser en termes de moyens humains, financiers et matériels, comment le gouvernement entend faire face à la situation dramatique des migrants. Oui, répondent la parole est à monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice. Le problème de la crise migratoire. Est un problème qu'il faut aborder avec beaucoup d'humilité. J'ai regardé l'évolution des chiffres. Dans votre département sur 2016, nous avons constaté une augmentation des demandes d'asile de plus 57 pourcent,, dont 786 était sous la procédure du au 1er semestre de cette année sur 1938 demandeurs d'asile 969 sont en procédure Dublin une augmentation de 50 alors nous avons décidé avec le président de la République, avec le 1er ministre. De mettre en place un plan qui nous permettent d'abord de pouvoir faire en sorte que. Les migrants qui arrivent aujourd'hui de Dublin, qui ont été déboutés du droit d'asile dans le pays où ils étaient et qui essayent aujourd'hui de venir en France puisse être traités en priorité, parce qu'autrement nous n'arriverons pas à faire face. Mais en même temps, nous voulons agir avec générosité et c'est pourquoi, sur un département comme le Pas-de-Calais nous avons fait en sorte que Sangatte la ne se reproduise plus, et c'est pour cela que nous venons d'ouvrir 200 d'accueil mais aussi de centres d'orientation.

avec Madame la ministre des solidarités, de la santé dans sa visite d'un centre d'hébergement d'urgence à Ivry, où il y a une grande implication de la Ville de Paris, de la municipalité d'Ivry d'un certain nombre d'associations dont Emmaüs et ceux dont les migrants ont besoin et les associations, il y a les les collectivités, c'est non pas de de moyens constants mais de moyens supplémentaires, parce que tout ne peut pas reposer sur le bénévolat, il faut que l'État sommeil et notamment au niveau des services publics, il y a des expériences qui fonctionnent, autant s'en servir et les multiplier pour la Cimade, pour 110000 demandeurs d'asile, ce sont plus de 30000 places nécessaires afin d'éviter toute mise à la rue, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant notre collègue Yannick et Vaugrenard pour le groupe socialiste et républicain pour 2 minutes. Merci monsieur le président, ma question s'adressait s'adresse toujours 1er ministre monsieur le 1er ministre vous avez annoncé une diminution de 5 euros par mois, du montant de l'aide personnalisée au logement et pour ses locataires touchant l'APL, ça n'est pas rien pourcent des des bénéficiaires ont des ressources inférieures au SMIC et plus de la moitié des ressources inférieures au seuil de pauvreté, voilà la triste réalité, cette mesure sur les appels est aveugle, elle frappe les plus pauvres, vous devez la supprimer chacun a intégré le fait que notre pays doit faire des économies afin que nos enfants et petits-enfants ne paient pas les pots cassés les pots cassés de l'irresponsabilité, mais Monsieur le 1er ministre pas de cette façon, pas comme cela auprès de ceux qui supportent déjà le calvaire des fins de mois difficiles pendant que d'autres pourront se satisfaire de voir leur impôt sur la fortune diminuer qui plus est, il y a dans ce projet une petite musique fort déplaisante, qui consiste à montrer du doigt, celles et ceux qui, dès lors qu'ils touchent les aides sociales seraient considérés comme des assistés, voire même des fraudeurs, nous vivons, mes chers collègues, curieusement, dans un monde où ceux qui gagnent 20000 euros par mois persuade ceux qui en gagne 10800 que tout va mal à cause de ceux qui vivent avec 535 euros et ça marche, hé bien moi je vous dis ça suffit. C'est en effet stigmatisant. De diminuer de 5 euros par mois, l'aide personnalisée au logement pour 6 millions 500 1000 ménages parmi les plus défavorisés, je vous suggère de prélever 0,0 7 pourcent sur le Patrimoine des 500 plus grosses fortunes de France ou encore 12 euros par mois sur les 10 pourcent des des revenus les plus riches, ce qui rapporterait strictement la même somme et serait beaucoup plus équitable, je vous demande solennellement, Monsieur le 1er Ministre revenez sur cette mesure parce qu'elle est injuste parce qu'elle touche aussi 800000 jeunes qui ont besoin d'être écoutés, d'être soutenu et non stigmatiser l'ensemble des associations caritatives et humanitaires, plaide pour sa suppression, je vous remercie, après m'avoir écouté de bien vouloir les entendre. Bon vous répond : la parole et au ministre de la cohésion des territoires Jacques Mézard, vous avez la parole. Sur le président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, Vaugrenard, je connais, monsieur le sénateur, Vaugrenard pour avoir été souvent assis dans cet hémicycle, votre souci de préserver nos concitoyens les plus fragiles, mais je vous dis très clairement aussi qu'il ne faut pas pousser la simplification trop loin, pourquoi le gouvernement a été amené à proposer avec regret cette mesure où, le savez aussi bien que moi, aussi bien que nous, c'est qu'il y avait donc dans le budget, une sous-budgétisation des APL, c'est la stricte réalité car vous aviez le gouvernement précédent et je le dis très clairement, avait prévu des mesures d'économies sur les APL qui n'ont pas été mis en place ce cas ce qu'a d'ailleurs, me semble-t-il reconnu, très loyalement l'ancien 1er ministre Manuel Valls je crois qu'il est nécessaire aussi de dire parce que ça a été un des soucis du Sénat ici en 2015 de demander par sa commission des finances, une enquête à la Cour des comptes sur le système des APL et à la suite de cela, il y a eu un rapport fait par le sénateur Dallier, de la même manière, à l'Assemblée nationale, il y a eu un rapport fait par votre camarade Monsieur Pupponi qui a conclu à quoi, à la nécessité de revoir ce système et de réaliser un certain nombre d'économies, y compris, y compris sur les allocations concernant le système des étudiants, donc ce que nous souhaitons parce que la réalité, elle est là, c'est constater les inégalités qui existent aujourd'hui dans le système, la complexité du système et je vous renvoie à la page 31 du rapport Madame facs qui est tout à fait révélateur à ce niveau-là, des efforts à faire pour rendre plus équitable effectivement les critères d'accès aux APL et de réaliser une politique du logement, qui nous permettent de faire d'aller vers une baisse des loyers et une relance de la construction, voilà la réalité, on peut pas éluder la réalité et le concret. Merci monsieur le ministre. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question concerne même pas que des sanctions américaines contre la Russie, en particulier en matière commerciale pour la France et pour l'Union européenne la semaine dernière, la Chambre des représentants américains a adopté de nouvelles sanctions, la grande, de la Russie, si le président Trump a la possibilité de sanctionner les entreprises qui travaillent sur des pipelines venant de Russie en limitant leur accès aux banques américaines et en les excluant des marchés publics américains, cela touche entreprises français Engie les allemands Uniper c'est Wintershall ou l'anglo-néerlandais Shell, merci, mes chers collègues qui travaillent sur le projet de gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne via la Baltique nous conduit de gaz en haut habitations sont remplis de gaz qui arrivent de Russie par tuyau et se remplit de gaz de schiste qui arrivent des États-Unis par bateau, notre première réaction devrait être d'arrêter d'acheter du gaz de schiste américain, c'est une compétition internationale États-Unis sont aujourd'hui largement excédentaire dans leur balance commerciale en matière de gaz, mais le problème est plus vaste cette décision américaine pose 2 problèmes : le 1er diplomatique, les décisions de sanctions contre la Russie, ont toujours été prises en concertation entre Zaz unies et l'Union européenne, ce n'est pas le cas cette fois-ci le second économique et commerciales, il est clair que l'impact sur les entreprises 17 heures énergétiques et en particulier gazier sera négative pour les entreprises européennes, la guerre commerciale dans ce domaine fait rage, cette situation pose le problème de la portée et extraterritorial des règles américaines qui coûte près de 20 milliards de dollars de pénalités aux entreprises européennes, selon le rapport de Pierre Lelouche et de Karine Berger sur ce sujet, notre propre commission européenne du Sénat, je vais retrouver tout

Vous avez la parole madame la mine. Monsieur le président Gbagbo, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Yves Pozzo di Borgo, comme vous l'avez indiqué le président Trump s'apprête à promulguer le projet de loi adopté largement par le Congrès américain, pourtant, de nouvelles sanctions contre la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, le recours à des sanctions est un outil de politique étrangère, auxquels nous ne sommes pas hostiles, le Conseil de sécurité des Nations unies a recours, l'Union européenne également, et en règle générale, nous examinons en concertation, les régimes de sanctions avec nos partenaires, en particulier au sein du G7 mais vous soulignez très justement le caractère particulier du projet de loi dont il est question, en particulier sa dimension extraterritoriale puisqu'il est, il rend possible de sanctionner des individus et des entreprises non américaines et notamment européennes en fonction de leurs activités qui ne sont pas liés avec les États-Unis, vous avez mentionné justement le rapport Lelouch Berger de l'Assemblée nationale, je pourrais rajouter le rapport bonne Carrère de cette haute assemblée qui dans les 2 cas, souligne les difficultés posées par les sanctions extraterritoriales et ouvre des pistes publiquement, nous avons indiqué que le caractère illicite au regard du droit international de ce de ces sanctions extraterritoriales, nous nous concertons d'abord avec l'administration américaine, Jean-Yves Le Drian a effectué une démarche auprès de Rex Tillerson pour marquer notre préoccupation Rex Tillerson a indiqué qu'il allait se concerter avec les alliés des États-Unis sur ce régime de sanctions plus largement, nous nous concertons avec nos partenaires de l'Union européenne, nous avons des outils qu'il s'agisse de mesures commerciales bien sûr de démarches diplomatiques, n'oublions pas aussi le règlement de 1996 qui avait été pris à la suite de la législation aux couleurs tonnes et qui permet de prendre des mesures de réciprocité en matière de sanctions commerciales, nous sommes donc mobilisés et nous soutenons les déclarations et les volontés d'action du président Junker je vous remercie. Merci, la parole est maintenant à notre collègue Patrick sièges pour le groupe, les républicains. Monsieur le président, ma chère collègue, ma question s'adresse à Monsieur le secrétaire d'État chargée du numérique si les collectivités se félicite que le sujet de l'aménagement numérique fasse partie des dossiers prioritaires du gouvernement s'interroge néanmoins sur d'éventuels changements d'orientation concernant bien sûr le calendrier mais aussi bien évidemment le budget aussi, il serait très utile dans un 1er temps de clarifier nettement les 2 échéances de 2020, d'une part celle qui consiste à rendre raccordables en fibre optique à la maison, l'ensemble des prises de la zone laissée à l'initiative privée et, d'autre part, la seconde échéance annoncée par le président de la République lors de la conférence des territoires qui a évoqué une bonne couverture haut et très haut débit pour tous il convient par ailleurs que les moyens nécessaires suivent pour confirmer l'échéance du plan France très haut débit en 2022, il faut en effet rassurer les collectivités qui doivent déposer dans les mois qui viennent, des dossiers de financement sur les 3,3 milliards d'euros d'autorisations de programmes, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste encore 250 millions d'euros inscrire finance pour assurer la cohésion des territoires, il est nécessaire que le gouvernement fixe un objectif conforme à celui de la Commission européenne soit un réseau permettant de livrer du 10 gigabits et des débit symétrique en 2025, c'est-à-dire en pratique en fibres jusqu'à l'abonné, cela signifie, selon les estimations de l'Agence du numérique de devoir inscrire 2 à virgule 5 à 2 milliards d'euros supplémentaires en autorisation de programme au moment où certains acteurs du secteur se déchaînent conquérir avec pour principal objectif de retarder le plus possible le déploiement du FTTH sur l'ensemble du territoire, il est impératif qu'une clarification vous apporter aussi Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous préciser l'échéancier nous rassurer sur les financements et enfin nous assurer que votre gouvernement préservera les investissements publics contre les attaques des opérateurs privés, je vous remercie.

et avec le ministre Maizar monsieur de Normandie et monsieur Griveau, ça a été notre première axes de travail, nous souhaitons trouver à la fois des solutions actives able rapidement et qui seront durables dans leurs effets, vous avez abordé 3 points le calendrier, la méthode, le financement, je répondrai à chacun sur le calendrier, un principe simple : nous ne changeons pas nous ne remettons pas en 15 les engagements passés, au contraire, nous allons plus vite, et c'était l'engagement du président de la République et concrètement qu'est-ce que ça veut dire sur 2020 sur 2020 du bon débit pour tous du monde des bitures plutôt, c'est pour cela, il va falloir s'engager à la fois sur l'accélération du réseau fixe sur l'accélération du réseau mobile, vous l'avez bien entendu 2020, ces 2 ans avant 2022 2022, sur lequel nous conservons l'engagement. 2022, sur lequel nous vous riez, certains parlent d'impatience numérique, les Français sont dans l'exaspération numérique, ne pas avoir le numérique aujourd'hui au quotidien, c'est être exclu, donc on ne peut pas rire de cela quand on annonce 2 ans d'avance sur leur engagement, nous devrions ici être tous ensemble mobiliser 2022. 2022, je répète, conservation de l'engagement du très haut débit pour tous et qui passera très majoritairement par le très haut débit, vous venez de parler d'un nouvel engagement qui est celui de 2025, il faut le rappeler, la société du gigabit, celle qui a été souhaité par la Commission européenne et qui veut dire près de 100 mégas pour les particuliers et 1 giga pour les équipements essentiels, les commerçants, les universités, les écoles, hé bien, cela reste l'objectif du gouvernement et nous irons jusqu'au bout sur la méthode, comment on fait pour changer ces dates, comment on fait pour aller plus vite, hé bien tout cela, il a fallu qu'on le fasse avec les acteurs et c'est pour ça que nous les avons réunis à plusieurs reprises avec 3 éléments majeurs redemander à chacun de ces aspects de ses acteurs, le respect de ses engagements et leur demander à chacun de présenter des gages pour la suite, puisque vous l'avez dit faut conclure mais il y a eu un problème sur la tenue des engagements améliorer accélérer les investissements et enfin l'innovation en s'ouvrant un nouveau mix technologique permis aujourd'hui par les nouvelles technologies enfin, sur le financement, et je le ferai au moins 10 secondes l'État s'est engagé et sur ses engagements, les collectivités peuvent faire confiance et enfin sur la suite,

Merci monsieur le président, Monsieur le 1er ministre vous êtes engagé à produire un effort budgétaire sur le quinquennat de 60 milliards d'euros lorsque le précédent gouvernement, est arrivé au pouvoir, les déficits s'est levé à 5,2 pourcent du du PIB au terme de ce quinquennat en ajoutant les correctifs de la Cour des comptes pour l'année 2017, que je ne remets pas en cause ici, il s'élève à 3,2 pourcent,, soit une baisse de 2 points du PIB environ 40 milliards d'euros j'ai avec monsieur dans le même temps, a eu une baisse de charges des entreprises de 40 milliards d'euros environ, financé pour moitié par des économies, ce qui fait 20 milliards d'euros, 40 milliards

commission des finances que les collectivités territoriales ont été amplement mise à contribution avec la diminution réalisé de leurs dépenses de 3 milliards d'euros en 2016 notamment, elles ont déjà donc prise la responsabilité, il faut savoir le dire, il faut aussi savoir le reconnaître monsieur le 1er ministre vous êtes en responsabilité, vous faites face à une situation des comptes publics, cela nous pouvons parfaitement l'accepter, ce qui pose problème au point de susciter un malaise jusque dans les rangs de la majorité, c'est la méthode, la méthode de la durable ou la méthode des baisses indifférenciées, par exemple, l'APL baisse de 46,5 millions de de budget sur la politique de la ville, sur la 2 tiers également et et les autres, mais tous les postes budgétaires à contribution, c'est une force le faire dans la méconnaissance des spécificités de chacun, c'est une injustice, je rappelle que le président de la République lui-même a souhaité mener la transformation des politiques publiques et appelé à mettre fin à cette vieille technique du rabot monsieur le 1er ministre donc je vous demande si ce n'est pas leur mettre en Côte, vos objectifs, c'est de changer la méthode et de mettre un terme à la politique du rabot et de prendre l'engagement solennel de préserver l'effort des territoires ruraux qui n'en peut plus et qui n'ont que trop contribuer au redressement des comptes merci. ce qui est sûr, c'est que nous devons mettre fin à l'idée que nous pouvons vivre indéfiniment en déficit est-ce qu'on imagine une entreprise est-ce qu'on imagine une famille qui, pendant plus de 40 ans vit en déficit

au gouvernement aujourd'hui 2400 euros par seconde, ce déficit se creuse 2200 milliards de dettes alors la méthode, évidemment, est très différent du gouvernement précédent, bien sûr, tout le monde a contribué mais pas en baisse de notation décidé uniformément par le gouvernement vis-à-vis des yeux locaux nous allons contractualiser avec nous allons discuter, ce sont, d'élus et le ministre d'État, Gérard Collomb, Jacques Mézard sur la demande du 1er ministre et du président de la République et moi-même, allant travailler avec l'ensemble des élus et des associations d'élus qui, effectivement, les collectivités locales puissent contribuer à l'effort des dépenses publiques, mais moins de façon moins importante que sous le quinquennat précédent propension puisque l'État va prendre la plus grande part de cette baisse de dépenses publiques aujourd'hui aujourd'hui, l'État n'a pas pris sa part totalement, il est vrai dans le gouvernement précédent sur la baisse des dépenses publiques et le budget que nous allons présenter est un budget qui sera à la fois sincère, nous allons ça séries et les dépenses, le Parlement pourra discuter des vrais inscription budgétaire dans ce budget, et nous allons pouvoir discuter d'un budget qui baissera qui baissera parce que nous ferons des vrais choix, ce sera pas l'eau coulera bon tout à fait raison madame la sénatrice quel concert de la politique, ce seront des choix et oui, nous avons choisi, à la demande du président de la République parce que les Français l'ont voulue, de baisser la fiscalité des entreprises parce que nous pensons que ce sont les entreprises qui créent l'emploi et c'est pas totalement l'accusation publique.

Monsieur le président, Mesdames et messieurs, féminisme et chers collègues, ma question s'adresse à Madame la Ministre, Jacqueline Gourault, Madame la Ministre, la conférence nationale des territoires en grande pompe devait rassurer les élus locaux depuis c'est exercice de communication, la réalité de vos annonces est venue les frapper de plein fouet la douche est froide, très froide, une baisse drastique des Budgets communaux se prépare dans aucune aux contreparties qui permet aux communes d'absorber le choc en plus de 11 milliards d'économies imposées aux Communes lors du précédent quinquennat ce sont 13 milliards d'euros qui vont leur être pris dans les 5 ans qui viennent, avec l'annulation par décret de 209 millions d'euros de crédits de paiement destiné à la politique des territoires et aux relations avec les collectivités locales, le coup est porté aux communes rurales avec la suppression de la dotation d'action parlementaire un marqueur de votre politique, les maires savent bien qu'ils ne pourront plus financer de très nombreux investissements avec la suppression de la taxe d'habitation, vous portez atteinte à l'autonomie financière des communes, enfin, le président de la République nous expliquer qu'il y aurait trop d'élus locaux, oubliant que 90 pourcent d'entre eux ne sont pas rémunérés alors qu'ils animent la cellule de base de notre démocratie. Quand arrêterez vous Madame la Ministre, la machine infernale qui creuse la fracture territoriale et prend les collectivités locales pour bouc-émissaire. Bonjour, répond : la parole est à Madame Jacqueline Gourault. Ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Intérieur pour 2 minutes. Merci monsieur le président. Mais, chers collègues, Madame la sénatrice, vous avez posé beaucoup de questions dans votre question, bien sûr, je vais y répondre, je vais essayer de répondre à toutes les questions d'abord commencer si vous voulez bien, par la diminution des élus locaux, le président de la République a rappelé qu'il dans les grands principes de la conférence des territoires que vous avez vous-même rappelé que, il y aura une liberté locale de laisser aux élus locaux pour s'organiser, exemple fusion département comme nouvelle etc et 9 mathématiquement bien sûr mathématiquement et engendrera bien sûr, la diminution du nombre d'élus locaux, il n'a jamais été question madame la sénatrice de diminuer le nord des élus locaux et de toucher au nombre de conseillers municipaux dans les communes, y compris les plus petites, je rappellerai au passage que dans la discussion de la loi notre, il avait été proposé ici même au Sénat qu'on envisage de diminuer, parfois, le nombre de conseillers municipaux devant la carence, il y avait parfois à faire des listes complètes, vous pourrez revérifier sur les finances locales Un des points le plus important de la conférence de territoires, c'est de passer un pacte comme vient de le rappeler, Gérald Harman avec les élus locaux, donc tout sera discuté dans cette conférence des territoires

à l'engagement que le président de la République a pris et je rappelle Madame pour terminer, que d'autres candidats à la présidence de la République ne disait pas 13 milliards d'économie, mais 20 milliards je vous remercie. Madame la ministre, il me semblait pourtant que nous parlions de même français la notation d'action parlementaire et là des c'est concrètement une maison de retraite une place du village, une cantine d'école, une église, son parvis, une maison de santé, ce sont des entreprises qui travaillent, des emplois, une économie locale vivante, vous étiez il y a quelques semaines encore, monsieur Maizar et vous-même membre de notre assemblée, et vous n'aviez pas de mots assez durs pour dénoncer les difficultés budgétaires que rencontrent les collectivités locales. notamment en milieu rural, il serait, à mon avis souhaitable et bienvenue que le ministre que vous êtes nous pas le sénateur. La parole est à Gilbert Roger. Pour le groupe socialiste et républicain. ma question s'adresse à Madame la Ministre des Sports, je me félicite de la qualité de la candidature de Paris pour l'organisation des Jeux olympiques 2 en 2024 notamment pour la Seine-Saint-Denis, qui accueillera 9 sites olympiques sur son territoire, je tiens à saluer la déclaration de candidature de Los-Angeles pour 2000 28 et c'est avec impatience que j'attends tout comme vous, la décision d'attribution du 13 septembre ce projet n'aurait pu voir le jour sans l'engagement du mouvement sportif qui a supporté avec conviction cette candidature, avec le soutien de l'État, initiée par le président Hollande est engagée par le président Macron et les collectivités territoriales concernées vocation a laissé un héritage durable au territoire en équipements sportifs en logements en infrastructures de transport aussi la Seine-Saint-Denis territoire jeune et dynamique doit se saisir de ce projet fédérateur pour transformer son image en requalifiant son territoire en créant des emplois, je souhaiterais aujourd'hui connaître les précisions du gouvernement en matière de sport tout d'abord, au-delà des grands équipements olympiques quels engagements le gouvernement pourrait-il prendre pour favoriser la l'accès à la pratique sportive de tous les enfants de Seine-Saint-Denis je pense en particulier aux plans piscine du conseil départemental alors que un enfant sur 2 en 6ème ne sait pas nager, je sais de quoi je parle, je suis maître nageur sauveteur en matière d'activité d'emploi: quelles mesures le gouvernement mettra-t-il en oeuvre pour favoriser l'accès des PME. à la commande publique face aux très grandes entreprises, il faut conclure généralisé les clauses d'insertion, voilà ma dernière question sociétés d'aménagement des sites olympiques pourront-elles participer à solide et au chargé de la livraison des sites à construire. Monsieur le président, Mesdames et messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, Gilbert Roger, l'attribution des Jeux à Paris en 2024 c'est un rêve depuis hier se rêve à la portée de nos mains le 13 septembre il devrait se réaliser 100 ans après les Jeux en guise de 1924 ça je serait l'incarnation de la France qui rayonne, merci à tous ceux qui se sont investis et qui ont porté cette candidature, vous l'avez dit merci à Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron année Hidalgo merci à cette France unie, qui défend les valeurs du sport, les valeurs humaines à cette France qui se rassemble derrière cette candidature et qui la porte d'une seule voix. Pour Paris et le Grand Paris, qui se concentreront une part importante d'acide et d'avis lâche pour une France entière avec des épreuves qui se dérouleront dans toute la France et un programme d'animation nationale qui sera menée sur le territoire d'ici à 2024 ça je nous offrirons une opportunité en faisant d'une du sport vecteur de nos politiques sportives publiques dans le domaine de la santé, l'éducation, la jeunesse, la culture, la lutte contre les discriminations en mettant ce projet fédérateur au service de la France et des Français, avec la création de 250000 emplois 4500 logements et un impact économique estimée à plus de 11 milliards d'euros, ils seront pour le territoire du nord du nord de Paris, un accélérateur exceptionnel de leur développement est un facteur d'innovation, les Jeux de 2024 seront la vitrine de l'excellence sportive française et offriront de nouveaux équipements nécessaires à la population tels qu'il a été prévu en concertation avec les élus locaux pour exemple effectivement le centre nautique qui va voir le jour en Seine-Saint-Denis où 50 pourcent des des enfants de moins de 11 ans ne savent pas nager aujourd'hui le 13 septembre prochain de nouvelles responsabilités de nouveaux défis, nous attendrons et les acteurs sportifs seront au coeur des performances attendues et c'est pour ça, c'est pourquoi je compte sur votre soutien merci.

Et quittera ses fonctions. Au terme d'une carrière de plus de 40 ans au service de notre institution. Aurait salué devant vous, mais sert collègues et au nom de tous les présidents qui m'ont précédé ici et qu'il a connu l'indéfectible loyauté dévouement de haute fonctionnaire à l'égard de notre assemblée, il fut notamment chef du service de la commission des lois, directeur de la science et enfin secrétaire général, je n'ai pas pu réaliser le nombre d'heures passées dans cette émission par Jean-Louis Hérin, mais aucun d'entre nous ne les atteindra jamais Monsieur le secrétaire général du Sénat tout l'hémicycle vraiment souhaite vous adresser ce message chaleureux, vous avez pu le le mesurer, vous arrêtez-vous demeurer un ardent défenseur, non seulement du Sénat mais tout autant d'un bicamérisme, indispensable à l'équilibre de nos institutions, à la place qui est la vôtre, vous avez constamment eu à coeur de musée à bâtir ce qui fait la spécificité sénatoriale l'attachement au pluralisme autant au contrôle et à la prospective, un débat qui sont ignorer les clivages privilégie chaque fois que cela est possible, la recherche de convergence dans un esprit de respect et d'écoute mutuelle, voilà pourquoi je ne voulais pas laisser passer cette séance sans vous saluer personnellement. A séance peut maintenant après 40 ans être levées. Et l'ordre du jour vous rappelle demain à ses heures, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour la confiance dans la vie politique, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi d'habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement. Du dialogue social et vous avez approuvé à l'unanimité, ma proposition vendredi après-midi à 15 heures la séance est levée.